L'augmentation s'élève à près de 750 millions d'euros en crédits de paiement, soit une progression de 4,3 % par rapport à 2022. Compte tenu de la masse salariale des universités, près de la moitié des crédits nouveaux sont consacrés à la mise en place pour 2023 de la compensation de la hausse du point d'indice pour les établissements d'enseignement publics. Il est à noter qu'aucune mesure de compensation n'aura été prise pour les mois de juillet à décembre 2022, pour lesquels les universités devront mobiliser leurs fonds propres.

Ces crédits sont essentiellement destinés aux dépenses de personnel, des mesures de revalorisation salariale et d'élargissement des voies de recrutement. Le PLF pour 2023 prévoit, en outre, la création de 413 emplois, dont 385 au titre de la LPR. Nous pouvons, je le pense, nous féliciter du renforcement des moyens ainsi consacrés aux universités, qui contribue à leur redonner des marges de manoeuvre et à limiter les tensions sur leur masse salariale.

Nous n'en sommes pour l'instant qu'à la phase de définition de cette expérimentation, mais je serai attentive à la négociation en cours entre le ministère et les universités. lequel devra s'exercer notre vigilance : du fait de la taille de leur patrimoine immobilier et des infrastructures de recherche qu'ils hébergent, y compris certains organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur sont particulièrement touchés par la crise énergétique. Le surcoût, en 2022, serait de 40 % à 50 % par rapport à 2021, soit près de 100 millions d'euros. de l'année 2023- et bien que l'évaluation des surcoûts potentiels soit un exercice délicat -, le ministère estime que le surcoût s'élèverait à 400 millions d'euros par rapport à 2022. Pour 2022, les universités devront mobiliser leurs fonds de roulement pour tenir compte de ces hausses. En 2023, elles bénéficieront du fonds de compensation du surcoût de l'énergie qui vient d'être voté par notre assemblée en projet de loi de finances rectificative. Si, sur le principe, cela semble un signal très positif pour les universités, seuls 150 millions d'euros de nouveaux crédits sont en réalité ouverts dans la loi de finances rectificative. les 125 millions complémentaires sont en partie financés sur les crédits dégagés par la baisse du nombre d'étudiants boursiers. Le constat de la vulnérabilité des établissements d'enseignement supérieur aux difficultés énergétiques me conduit à aborder les enjeux cruciaux d'investissement dans le patrimoine immobilier universitaire.

« Vie étudiante » avaient enregistré une hausse très importante ; le projet de loi de finances pour 2023 prévoit leur stabilisation. Le montant des bourses sur critères sociaux a été revalorisé de 4 % à la rentrée 2022 afin de tenir compte de l'inflation. Le coût de cette mesure est chiffré à 85,1 millions d'euros en 2023, mais les crédits dédiés restent identiques à ceux qui étaient prévus l'année dernière, du fait de la baisse attendue du nombre d'étudiants En outre, cette revalorisation ne permettra pas de couvrir l'érosion du pouvoir d'achat découlant de l'inflation constatée en 2022 et prévue en 2023. parallèle, la subvention versée au réseau des oeuvres universitaires progressera de 35,6 millions d'euros par rapport à 2022, pour financer notamment la prolongation du ticket U à un euro pour les étudiants boursiers et le gel des loyers dans les résidences étudiantes.

Là encore, je soulèverai un point d'attention : la hausse du coût des denrées alimentaires pourrait engendrer un effet ciseau, le nombre de repas servis augmentant parallèlement au renchérissement du prix des matières premières. et scolaires (Cnous) font état d'une possible hausse des effets directs du repas à un euro pour la fin de l'année, le coût total étant de l'ordre de 50 millions d'euros- nous devrons y être très attentifs, madame la ministre.

supplémentaires sont ainsi prévus pour 2023 afin de respecter les engagements qui ont été pris dans le cadre de la loi de programmation. Nous pouvons, me semble-t-il, nous en féliciter.

découlaient d'un tel choix. Il est vrai que l'inflation était alors très faible, ce que n'avait pas manqué de faire valoir le Gouvernement. Dans la situation actuelle, la loi de programmation aura surtout protégé la mission « Recherche et enseignement supérieur » d'une érosion de ses moyens liée à l'inflation. La clause de revoyure figurant dans la loi de programmation prévoyait une actualisation de la programmation au moins tous les trois ans. J'espère, madame la ministre, que cette occasion sera saisie en 2023 et que nous pourrons en rediscuter. Par ailleurs, de nombreuses infrastructures de recherche sont très consommatrices d'électricité et seront par conséquent très affectées par la hausse des coûts énergétiques en 2023. Je souligne notamment les difficultés auxquelles

mise en oeuvre de la LPR expliquent le reste de l'augmentation enregistrée en 2023. Celle-ci a trait notamment à l'amélioration des carrières dans la recherche, à la rémunération des doctorants et à l'augmentation des moyens alloués aux laboratoires et aux grandes infrastructures de recherche nationales et internationales. Il est indéniable que ces moyens nouveaux vont redonner des marges de manoeuvre aux organismes de recherche. Alors que la subvention pour charges de service public versée aux opérateurs subissait année après année une lente érosion, le budget pour 2023 confirme l'inversion de tendance qui avait pu être espérée en 2022.

pour bien régler la voilure, il fallait 1 milliard d'euros et 25 % de taux de succès- on y est presque. De manière générale, le redressement financier de l'ANR constitue un signal très encourageant pour nos chercheurs. Il me semble que nous devons être attentifs aux enjeux d'articulation avec les appels à projets européens,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon propos sera essentiellement centré sur les crédits de la mission interministérielle pour la recherche et l'enseignement supérieur (Mires) entrant dans le périmètre de la commission des affaires économiques. Les crédits de la mission sont en hausse, conformément à la trajectoire budgétaire conformément à la trajectoire budgétaire et à la trajectoire d'emploi prévues par la LPR. Depuis deux ans, j'ai pris l'habitude de vous dire que je n'auditionne que des gens heureux. Cette année, je trouve les gens heureux, mais soucieux ! En effet, ce projet de loi de finances est marqué par la hausse des prix et des coûts de l'énergie, dont les répercussions sont, me semble-t-il, sous-estimées. En 2020, le Sénat avait attiré l'attention du Gouvernement sur le fait que la trajectoire budgétaire prévue par la LPR était calculée en euros courants et non en euros constants, c'est-à-dire sans prise en compte de l'inflation ; il nous avait été répondu que l'inflation était une donnée économique qui appartenait au passé. Force est de constater que la situation que nous vivons nous donne raison. Les écarts prévisionnels de trajectoire sont importants : au moins 50 millions d'euros en 2023 et jusqu'à 400 millions d'euros en 2027 si aucune mesure n'est prise. Les budgets des opérateurs de recherche sont d'ores et déjà touchés par l'inflation et par la hausse des coûts de l'énergie. Ces surcoûts

Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds demeurent floues. Je me permets d'insister sur deux points : d'une part, l'ensemble des grands organismes de recherche doivent pouvoir bénéficier de ce fonds ; d'autre part, les versements doivent s'effectuer au prorata des surcoûts énergétiques et non de façon forfaitaire par établissement. Les budgets sont également touchés par le dégel du point d'indice des fonctionnaires décidé au mois de juillet 2022. Si des compensations sont prévues en 2023, ce n'est pas le cas pour le second semestre 2022.

de budget prévues par la LPR doivent avant tout permettre de soutenir nos activités de recherche et de porter notre effort national de recherche à 3 du PIB, alors que nous stagnons depuis plusieurs années à seulement 2,2 % du PIB. La clause de revoyure de la LPR prévue en 2023 devrait être

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur les crédits du programme « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Recherche et enseignement supérieur

française. La situation actuelle est marquée par une inflation des prix de l'énergie- cela a été dit -, exposant nos opérateurs à l'explosion des factures énergétiques. Malheureusement, il est à craindre que l'augmentation des crédits ne permette pas de compenser les surcoûts.

Des opérateurs tels que le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), IFP Énergies nouvelles ou encore l'université Gustave-Eiffel sont, dans leurs domaines respectifs, de véritables pionniers, que dis-je, de véritables pépites. En témoigne le nombre important de brevets déposés par ces acteurs de pointe, traduisant une véritable reconnaissance de l'expertise française et démontrant une capacité à investir de nouveaux sujets de recherche. De même, des projets déployés à l'échelle européenne ou internationale mettent en lumière la maturité de la recherche française ; je pense ici à l'implication de la filière aéronautique française dans la création d'avions de ligne bas-carbone à l'horizon 2023. Perpétuer dans la durée le soutien accordé aux opérateurs nous permettra de répondre à un double enjeu.

Le second enjeu est d'éclairer les choix des décideurs afin de lutter efficacement contre le changement climatique et de garantir une maîtrise des risques environnementaux, industriels et nucléaires.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, tout comme mon collègue rapporteur spécial, j'exprime ma satisfaction de voir le budget de la recherche poursuivre son augmentation en 2023, sous l'effet du déploiement de la loi de programmation de la recherche. Sa troisième annuité permettra d'abonder de 400 millions d'euros supplémentaires la Mires, évolution respectueuse de la programmation que nous avons votée, ce qui mérite d'être salué. Je me félicite aussi que vous ayez pris l'initiative, madame la ministre, d'aller plus loin que la LPR quand la situation le nécessitait. C'est ainsi le cas pour la revalorisation de la rémunération des doctorants, que vous avez décidé d'étendre aux contrats en cours. Il s'agit là d'un signal très positif pour nos doctorants 2023 sera aussi la troisième année de montée en charge financière de l'Agence nationale de la recherche, dont nous observons d'ores et déjà les retombées positives pour nos chercheurs : le taux de sélection aux appels à projets atteint aujourd'hui 23,5 %, contre 17 % en 2020, et le taux de préciput s'élève à 28,5 %, pour un montant de 200 millions d'euros. Ces premiers résultats sont très prometteurs, mais ils se heurtent malheureusement à la réalité économique. Le rapporteur spécial l'a rappelé, le Sénat avait alerté sur le manque de crédibilité de la trajectoire budgétaire sur dix ans, car elle ne tenait pas compte de l'inflation. Deux ans plus tard, le choc inflationniste que connaît notre pays est tel que l'effort budgétaire de la LPR est largement absorbé. Pour notre commission, il est donc indispensable que la clause de revoyure prévue en 2023 soit mise à profit pour rectifier la trajectoire, d'une part, en ramenant sa durée à sept ans, comme nous l'avions demandé initialement, afin d'atténuer les risques liés aux aléas macroéconomiques ; d'autre part, en augmentant l'intensité des prochaines annuités, afin de créer les conditions du réinvestissement massif dont notre recherche a besoin. Devant notre commission, madame la ministre, vous vous êtes engagée à nous transmettre d'ici à la fin de l'année un premier bilan de la mise en oeuvre de la LPR et, sur cette base, à examiner la faisabilité d'une accélération de la trajectoire. Je compte donc sur votre détermination, mais aussi sur notre mobilisation, mes chers collègues, pour faire de la clause de revoyure en 2023 un rendez-vous constructif et ambitieux, qui puisse trouver sa traduction budgétaire dans le projet de loi de finances pour 2024. Ce rendez-vous sera d'autant plus attendu que l'année 2023 suscite une forte inquiétude chez les opérateurs de recherche, pris à la gorge par les surcoûts énergétiques. Est-il besoin de rappeler que de nombreuses infrastructures de recherche sont très consommatrices d'énergie et que l'activité expérimentale ne peut être brutalement interrompue ? Vous avez réussi, madame la ministre- et je vous en félicite -, à obtenir de Bercy le déblocage d'un fonds exceptionnel de soutien, dont 55 millions d'euros iront aux organismes de recherche, qui devront aussi mobiliser leurs ressources propres. Espérons que ces fonds permettront à nos opérateurs de recherche de ne pas basculer dans le rouge Je conclurai en mettant un rapide coup de projecteur sur un sujet qui me tient très à coeur, la culture scientifique. La mesure du « 1 % ANR » de la LPR a eu un véritable effet catalyseur : loin d'être une simple source de financement, elle a créé un engouement, une dynamique, dont je me réjouis. De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour : le lancement d'appels à projets ciblés sur la culture scientifique, la création de prix récompensant les chercheurs engagés dans ce domaine, des campagnes de labellisation des sites universitaires accueillant des initiatives « culture scientifique ». Sous le

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je partage la satisfaction générale de constater l'augmentation de près de 750 millions d'euros des moyens consacrés à l'enseignement supérieur. La compensation de l'augmentation du point d'indice était évidemment très attendue des établissements, qui n'y ont pas eu droit en 2022 et qui, en conséquence, devront financer une demi-année de hausse sur leurs fonds propres. Ce surcoût de masse salariale vient s'ajouter au glissement vieillesse technicité (GVT), toujours non compensé à ce jour. Les établissements d'enseignement supérieur nous disent par ailleurs leur forte inquiétude face à l'ampleur des surcoûts énergétiques. Le déblocage d'un fonds exceptionnel doté de 275 millions d'euros est accueilli avec soulagement par les intéressés, mais suscite des interrogations. Madame la ministre,

Depuis que je suis rapporteur pour avis, je plaide pour le lancement d'un grand plan d'investissement destiné à la rénovation du parc immobilier universitaire, connu pour être très vaste, vieillissant, en partie vétuste et énergivore. La crise énergétique que nous subissons rend plus que jamais nécessaire une réflexion de fond sur la quantité et la qualité du bâti universitaire au regard des récentes évolutions pédagogiques et sociétales, l'avenir consistant sans doute en « moins de mètres carrés » pour « mieux de mètres carrés Durant la crise sanitaire, quand l'urgence était de relancer rapidement l'économie française, le Gouvernement a fait le choix de passer par la méthode de l'appel à projets pour encourager la rénovation énergétique dans Cette initiative a certes permis de donner une véritable impulsion, mais, compte tenu du retard accumulé ces dernières décennies et de l'ampleur des besoins d'investissement- évalués à 7 milliards d'euros par votre ministère, mais à plus du double par France Universités -, un changement d'échelle est indispensable. Je conclurai en tirant la sonnette d'alarme quant au financement de l'activité de restauration des Crous. Si, en 2022, la rentrée s'est déroulée dans un climat beaucoup plus serein que les années précédentes, les restaurants universitaires sont confrontés à une tension croissante. En deux ans, leur activité a augmenté, selon selon les sites, de 20 % à 40 %, sous l'effet de plusieurs facteurs : attractivité du repas à un euro, fidélisation de nouveaux étudiants, contexte inflationniste et conséquences de la loi pour Je m'étonne qu'il n'y ait aucun lien entre le volume de repas fournis et le niveau de la subvention versée au réseau, laquelle stagne depuis plusieurs années. Il est sans doute temps d'ouvrir ce chantier d'une remise à plat du financement de la restauration universitaire. Sous le bénéfice de ces observations et malgré ces quelques réserves, la commission de la culture a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits de l'enseignement supérieur pour 2023. Dans la suite

c'est très bien. Parlons-en ! Au sein des grandes écoles, la diversité sociale n'a pas progressé en dix ans. Si l'on devait brosser le portrait de leurs étudiants, on pourrait dire que leurs parents sont issus des catégories socioprofessionnelles supérieures et que, le plus souvent,

et commerciale générale sont privées, les frais annuels y dépassant en moyenne les 5 000 euros. Il existe aussi des officines privées, auxquelles les étudiants ont recours en parallèle de leurs enseignements, qui peuvent être très coûteuses et qui les aident à préparer les travaux dirigés et les examens.

L'enseignement public doit être la voie d'excellence. Tel est le cas pour les filières scientifique et littéraire ; il faut qu'il en aille de même dans toutes les disciplines. Le secteur du jeu vidéo, par exemple, dispose d'une seule formation supérieure publique, alors qu'il est en plein développement, propose des recrutements et constitue un domaine d'excellence pour la France. Les déterminants non académiques de la réussite ne doivent pas représenter un obstacle et le mérite doit demeurer un ascenseur social. La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants avait prévu que soit retenu, dans le cadre de la procédure Parcoursup, un taux minimal de bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée,

30 % jusqu'en 2025. Nous devons être plus ambitieux ! Je salue les mesures prises par le Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat des étudiants, comme le gel de l'indexation des loyers en résidence universitaire, la revalorisation de 4 % du montant des bourses sur critères sociaux et le maintien du repas

soit 25 millions d'euros de plus que l'année dernière. Il est important que la CVEC ne devienne pas un simple levier d'intervention face aux crises sanitaires et énergétiques, mais qu'elle favorise chez les étudiants, conformément à l'intention du législateur, la pratique sportive et l'accès à l'art et à la culture, c'est-à-dire au bien-être et à l'épanouissement. L'activité physique étant un important facteur d'épanouissement physique et psychique, je me réjouis de l'extension du Pass'Sport à 800 000 étudiants boursiers depuis la rentrée 2022.

La recherche, elle, n'a pas non plus été hermétique à ces épreuves. La question de la performance de la recherche étant posée au grand jour, l'occasion a été donnée de rappeler combien, dans certains secteurs, notre pays s'était endormi. C'est dans un tel contexte que nous avions examiné, à partir des travaux de notre collègue Laure Darcos, le projet de loi de programmation de la recherche. tant le budget de l'enseignement supérieur que celui de la recherche : manque de financements pour les revalorisations salariales ; manque d'investissements pour rattraper notre décrochage dans le domaine de la recherche ; manque de financements pour rénover les bâtiments universitaires vieillissants ; manque de financements, enfin, pour parer aux effets de l'inflation. Qu'en est-il dans le cadre de ce projet de budget pour 2023 ? Avons-nous progressé ? Allons-nous progresser ? Indéniablement, oui, puisque les crédits augmentent substantiellement : +1 milliard d'euros par rapport à 2022. Madame la ministre, je salue l'ambition forte que vous défendez et les résultats concrets s'articule autour de trois priorités, que vous avez rappelées : compensation pérenne de la revalorisation du point d'indice ; poursuite de la trajectoire de la LPR ; mesures nouvelles en faveur de la vie étudiante ou reconduction de mesures exceptionnelles mises en oeuvre depuis la crise sanitaire. Les moyens augmentent, des efforts significatifs sont réalisés afin de répondre à l'urgence que connaissent ces secteurs stratégiques pour l'avenir de notre pays. Dans le contexte d'inflation et de crise énergétique que nous connaissons, ces hausses de crédits permettent de tenir les objectifs

afin que les augmentations de moyens se traduisent réellement par un « choc d'investissements » et ne servent pas seulement à faire face à l'inflation. Le cas de la réhabilitation du patrimoine universitaire est parlant. Votre ministère évalue le besoin à 7 milliards d'euros, dont 75 % devraient être consacrés à la transition énergétique. L'appel à projets de 2020 avait permis de lancer certaines opérations, mais avait également exhibé l'ampleur des besoins. Le ministère continue donc d'accumuler du retard.

La revalorisation des contrats des doctorants, initialement réservée aux nouveaux entrants et que vous avez décidé d'étendre, ce qui est une bonne chose, ne doit pas occulter le besoin d'un travail de fond sur l'attractivité de la recherche. Les conclusions de notre collègue rapporteure pour avis Laure Darcos, qui relève que les postes créés par la LPR n'ont pas tous été pourvus, nous invitent également à une très grande vigilance. Madame la ministre, comme mes collègues du groupe Les Républicains, je voterai les crédits de cette mission. Je salue votre volontarisme pour défendre l'enseignement supérieur et la recherche. Toutefois, je vous exhorte à ne pas perdre de vue menées en ce domaine : mieux former les étudiants, mieux les orienter, lutter contre des taux d'échec qui restent importants. Voilà pourquoi je vous invite à vous rapprocher

Nous le disions voilà peu, à l'occasion d'un débat organisé par nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste : cette articulation ne fonctionne pas. L'enseignement supérieur n'a pas pris réellement la mesure du nouveau baccalauréat et cette non-prise en compte génère et nourrit l'échec de la réforme du lycée. Les attendus de l'enseignement supérieur ne peuvent plus ignorer le souci de donner plus de liberté et de choix aux lycéens et, par leur spécialisation progressive, de les aider à se muer peu à peu en étudiants. Les formations supérieures qui privilégient le tronc commun, celles qui, par leurs attendus, cherchent à reconstituer l'ancienne voie S, rendent un bien mauvais service à la réforme du lycée, et même au pays. Faire de l'orientation des lycéens et des étudiants une grande cause nationale, voilà ce qui manque à votre projet de budget comme à celui de votre collègue Pap Ndiaye. me semble pourtant indispensable de mettre en chantier ce lien lycée-licence, si souvent évoqué. Le nouveau baccalauréat aurait dû être l'occasion d'une réflexion de fond sur la mue progressive d'un lycéen en étudiant. Parce que l'instauration de Parcoursup dans l'urgence et la réforme du lycée ont été conçues en silo et selon un calendrier inversé, nous nous retrouvons dans la même situation qu'en 2017. L'articulation lycée-licence reste à construire. Votre projet de budget, par ailleurs volontariste, ne dessine pour autant aucune priorité en la matière. C'est dommage ! Résultat, les angoisses des futurs étudiants s'amplifient,

pourtant pas l'outil qui est en cause, même s'il doit être amélioré, ni la philosophie du nouveau baccalauréat, même si bien des calages restent à faire- on l'a vu pour l'enseignement des mathématiques. C'est la prise en compte de l'esprit et de l'organisation du nouveau baccalauréat

Cependant, près de la moitié des nouveaux crédits sont consacrés à la compensation de la hausse du point d'indice : on parle de 364 millions d'euros budgétés pour 2023. Comme l'a très bien expliqué Vanina Paoli-Gagin, rapporteur spécial de la commission des finances, l'ensemble des engagements inscrits dans la loi de programmation de la recherche sont respectés. Je m'inquiète en revanche de l'insuffisante prise en compte de la rénovation du parc immobilier universitaire dans les crédits alloués. D'après le ministère, le surcoût énergétique devrait s'élever à 400 millions d'euros. Ni la fermeture des universités quelques semaines supplémentaires ni la généralisation des cours en distanciel pour contrebalancer la hausse des coûts de l'énergie ne seront des solutions satisfaisantes. Le groupe Les Indépendants appelle donc à un investissement de grande ampleur en faveur de la rénovation énergétique de l'immobilier universitaire. universitaire. Les crédits consacrés à la vie étudiante augmentent de 1,5 %, à hauteur de 3,13 milliards d'euros en crédits de paiement. Le montant des bourses sur critères sociaux a été revalorisé de 4 % à la rentrée de 2022 pour tenir compte de l'inflation est extrêmement important de ne pas laisser les étudiants dans la précarité. Les repas à un euro, qui ont été distribués à plus de 430 000 étudiants boursiers lors de l'année scolaire dernière, sont maintenus.

de la mission, il augmente de 824 millions d'euros en crédits de paiement, atteignant 12,77 milliards d'euros. Notre groupe salue cette hausse qui est autant un choix qu'une nécessité. La stratégie française en faveur de ses chercheurs et de son industrie spatiale est déterminante pour rester en pointe. Soutenir la recherche est un enjeu de souveraineté essentiel dans la perspective

En revanche, la hausse des coûts n'a pas été prise en compte dans l'octroi des crédits, ce qui doit nous alerter au regard de l'actuelle tendance inflationniste. La forte hausse des crédits alloués à la recherche spatiale est une très bonne nouvelle. La Chine et les États-Unis investissent massivement dans l'espace et nous devons faire de même si nous voulons rester dans la course. Le montant global de ces crédits serait de 1,7 milliard d'euros pour 2023, soit une hausse de 74 millions d'euros à périmètre constant.

le retard du projet Ariane 6. Ce retard est d'autant plus dommageable qu'il fragilise la souveraineté européenne en matière de politique spatiale ; ce n'est pas l'élu toulousain que je suis qui restera insensible à ce

Premièrement, le budget pour 2023 se révèle conforme à la LPR et suit la trajectoire qui avait été définie, pour la recherche comme pour l'enseignement supérieur. Deuxièmement, l'État se doit de doter les enseignants des moyens nécessaires ; à cet égard, la hausse globale de la rémunération de 6 % va dans le bon sens. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants accueille favorablement ces crédits et les votera.

L'augmentation des moyens de l'ANR est une bonne nouvelle pour les futurs lauréats des appels à projets. Nous réitérons toutefois notre inquiétude concernant la place accordée aux financements par appels à projets : nous l'avons dit, s'ils constituent de bons compléments des financements récurrents,

Pour paraphraser un ancien Président de la République, nos forêts brûlent et nous contemplons les étoiles. Veillons à ne pas en faire notre maxime d'action

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

des mesures indemnitaires : revalorisations statutaires des personnels de recherche, repyramidage des maîtres de conférences et des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation, à hauteur de 75 millions d'euros.

cette mesure représente un effort financier de plus de 85 millions d'euros en 2023. Le Gouvernement a en outre annoncé le lancement d'une grande concertation préalable à une réforme des bourses sur critères sociaux.

Le réseau des oeuvres universitaires se voit doté d'une subvention pour charges de service public en hausse de 35,5 millions d'euros par rapport à 2022. Des créations de postes se traduisant par un schéma d'emploi de 40 ETP

de vous remercier

Mais cette bienveillance a ses limites, compte tenu des urgences auxquelles font face nos universités, l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur, les chercheurs et nos étudiants. La première de ces urgences, c'est la flambée des prix de l'énergie. Quelle ne fut pas notre stupeur, à la rentrée dernière, lorsque plusieurs présidents d'université ont annoncé envisager une fermeture temporaire de leurs établissements au coeur de l'hiver, par crainte de ne pouvoir faire face aux surcoûts liés à la hausse des prix de l'énergie ! ! Le souvenir douloureux des cours en distanciel, des enseignements tronqués, des difficultés d'accès aux ressources et de l'isolement grandissant de chacun a ressurgi.

Le parc universitaire représente 20 % du patrimoine immobilier de l'État, mais près d'un tiers de ces bâtiments sont des passoires énergétiques ! Nous proposerons, au cours de la discussion, des amendements tendant à remédier Deuxième urgence : le manque de moyens réels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Certes, le budget du ministère est en hausse et la trajectoire prévue dans la loi de programmation de la recherche est en apparence respectée. Vous pouvez vous prévaloir, madame la ministre, d'une hausse globale de 5 % des crédits alloués à la mission « Recherche et enseignement supérieur », qui passent de 29,07 milliards à 30,61 milliards d'euros. Mais que reste-t-il réellement de cette hausse une fois prise en compte l'inflation galopante- elle frôle les 6 % ? Dans les faits, les moyens baissent. baissent. Aux effets de l'inflation et aux surcoûts liés à l'énergie, il faut ajouter les non-compensations du glissement vieillesse technicité et de la hausse du point d'indice. Si la hausse du point d'indice de 3,5 %, soit un taux inférieur à celui de l'inflation, est bien compensée pour 2023, elle ne l'a été qu'à moitié pour 2022.

Pis, ces inégalités vont en se renforçant, y compris entre les sexes. Selon une récente note de l'Institut des politiques publiques, les étudiantes sont sous-représentées dans les filières et disciplines les plus coûteuses.

Comment peut-on étudier sereinement quand on vit dans un logement exigu, souvent loué à un prix exorbitant, quand la fac se trouve à plus d'une heure de transport, quand on doit faire appel aux banques alimentaires pour manger à sa faim ? Dans ces conditions, comment faire face à la charge de travail quotidienne à la fac, au stress des examens et à la pression de devoir trouver un emploi au sortir de l'université ?

il est apparu très clairement que la hausse de 4 % des bourses sur critères sociaux, votée à l'été, serait totalement insuffisante. Certes, madame la ministre, la concertation que vous avez lancée sur une réforme des bourses est bienvenue, mais notre jeunesse ne peut attendre : l'urgence est là ! Nous proposerons par conséquent plusieurs amendements visant à pallier le manque de moyens alloués à la vie étudiante. d'abord le retour du ticket-restaurant universitaire à un euro pour l'ensemble des étudiants. Il est indispensable de rétablir cette aide quotidienne pour tous les étudiants précaires qui ne bénéficient ni d'une bourse,

Alors que les deux années de covid-19 ont laissé des traces pérennes chez les jeunes et que la pression toujours plus grande à laquelle ils sont soumis met à mal leur santé mentale, le manque de psychologues sur les campus se fait aussi cruellement sentir. Nous sommes toutefois bien conscients que ces quelques amendements visant à lutter contre la précarité étudiante,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France délaisse ses universités. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner quelques chiffres. Depuis dix ans, la dépense moyenne par élève a augmenté de 1,5 % par an dans le premier degré et de 1,2 % par an dans le second degré. Cette progression continue s'explique par la conjonction de la stabilité des moyens budgétaires et de la baisse des effectifs. Le processus est inverse dans les universités, qui ont dû accueillir durant la même période un demi-million d'étudiants supplémentaires à budget constant. Ainsi la dépense moyenne par étudiant a-t-elle baissé en moyenne de 1,4 % tous les ans depuis 2014. En revanche, elle est restée stable pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, qui ont

Il serait très préjudiciable à la qualité pédagogique des enseignements et à la réussite des étudiants que ces apories budgétaires aient finalement pour conséquences de nouvelles régressions des taux d'encadrement. Les universités, comme les collectivités, sont en quelque sorte placées sous la curatelle budgétaire de l'État pour assurer leurs missions de service public. Cette dépendance accrue est la conséquence du conflit entre la hausse de la démographie, le principe constitutionnel d'égalité d'accès des étudiants à l'université et l'inadéquation des dotations de l'État. Cette « striction » malthusienne induit une recentralisation de la maîtrise budgétaire au profit des administrations et, à terme, la fin de l'autonomie des universités.

À l'origine de cette carence organisée, il y a le calcul budgétaire de Bercy, qui considère que la baisse attendue de la démographie estudiantine redonnera des marges budgétaires aux établissements. Je ne partage pas cette projection stratégique, car elle ignore les objectifs d'une baisse du taux d'échec en licence et d'une hausse du taux de poursuite des études universitaires.

Le ministère des solidarités estime que 40 % des étudiants qui vivent seuls sont en situation de pauvreté. Pendant la crise sanitaire, ils avaient été privés de leur emploi ; désormais, ils subissent avec une grande violence l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie.

Ainsi est-il absurde de concentrer l'offre d'études supérieures dans les métropoles, alors que ces villes sont soumises à une pression sans cesse accrue en matière de logement. Dans de nombreuses régions, le premier poste de dépense des étudiants, c'est le logement

Les universités et les étudiants ne peuvent plus être systématiquement ignorés des politiques sociales. Ils doivent être placés au coeur des ambitions de l'État. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Pour commencer, j'évoquerai la précarité étudiante. Après deux années de pandémie mondiale, la rentrée 2022 a été synonyme de retour à la normale pour la majorité des étudiants.

donc, un grand nombre d'étudiants, ne s'arrêtera pas avec l'hiver. Des dispositifs sont-ils prévus en vue du printemps ? Si ce fonds répond à une situation d'urgence, il ne constitue pas une solution pérenne. La situation des Crous, qui ont été très sollicités durant la crise sanitaire, continue de s'améliorer et les crédits qui leur sont alloués sont en constante augmentation. Cependant, la hausse des prix des denrées alimentaires pourrait engendrer un déséquilibre.

Comme le covid-19 a précipité la digitalisation, la crise énergétique rend la transition environnementale encore plus urgente. Alors qu'il est impératif de lancer un plan massif de rénovation de ce patrimoine, la dotation budgétaire consacrée à l'immobilier universitaire Cet effort ponctuel demeure insuffisant et ne permettra pas à la France d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés en matière de transition énergétique. Cette réflexion doit aussi englober les laboratoires, dont les matériels scientifiques sont bien plus énergivores que le chauffage des amphithéâtres. Ainsi Esiee Paris, école d'ingénieurs comptant parmi les membres de l'université expérimentale Gustave-Eiffel, possède-t-elle une salle blanche qui concentre à elle seule plus ou moins la moitié des dépenses énergétiques de l'école. Les crédits des programmes du volet « Recherche » de la mission devraient atteindre, en 2023, 12,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution résulte essentiellement de l'ajout d'une enveloppe de 330 millions d'euros allouée aux organismes de recherche du programme 172, ainsi que de la forte hausse des crédits consacrés à la recherche spatiale.

Cependant, cette trajectoire ne prend pas en compte l'inflation, ce que nous avions déjà regretté à l'époque, et ce que nous continuons de dénoncer. La LPR prévoyait une actualisation de la programmation tous les trois ans. devrions donc, en 2023, rediscuter de l'ensemble de ces sujets. Nous espérons que le Parlement sera associé à l'ensemble de cette réflexion. D'ici là, madame la ministre, vous pouvez être assurée que nous soutenons les efforts consentis par le Gouvernement : nous voterons en faveur de ces crédits.

On peut également relever la hausse des crédits demandés pour le programme 150, qui permet de porter à 14,9 milliards d'euros pour 2023 le budget relatif aux formations supérieures et à la recherche universitaire. Toutefois, si cette hausse globale des crédits nous semble aller dans le bon sens, elle ne saurait masquer les graves difficultés auxquelles sont confrontés les établissements de l'enseignement supérieur, leur personnel et leurs étudiants.

Les universités sont particulièrement touchées, car elles hébergent une grande majorité des laboratoires et infrastructures très énergivores. Déjà, la facture pour l'année 2022 a fait apparaître un surcoût estimé à plus de 100 millions d'euros par rapport à 2021.

Le calcul est simple : la hausse des prix de l'énergie va entraîner pour nos établissements un surcoût de plus de 500 millions d'euros pour les années 2022 et 2023. Pour y parer,

certains chantiers de démolition sont freinés. Il est donc urgent d'agir, à court terme et à long terme, afin de réhabiliter le parc immobilier universitaire. C'est indispensable si nous voulons que nos universités atteignent l'objectif de réduction de 40 % de leur consommation

Mais les moyens mis en oeuvre ne nous paraissent pas suffisants, car le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter, année après année. L'évolution de la dépense moyenne par étudiant continue de baisser. Le rapport 2023 sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures indique même que, de 2013 à 2021, le coût moyen par étudiant à l'université a baissé de presque 15 %.

vous avez décidé d'augmenter les bourses de 4 %, vous gelez les loyers des résidences universitaires et vous étendez le Pass'Sport aux étudiants boursiers. Une inquiétude demeure cependant concernant les restaurants universitaires, de plus en plus prisés des étudiants en raison de leur faible coût. Si vous avez décidé de maintenir le repas

À ce sujet, on ne peut que s'étonner que la subvention pour charges de service public du réseau (SCSP) soit stabilisée à 300 millions d'euros au lieu d'être revue à la hausse, alors que l'activité de restauration s'accroît considérablement depuis la crise sanitaire, que le réseau poursuit son développement et qu'il se voit confier des missions supplémentaires d'accompagnement social des étudiants. Madame la ministre, nous ne comprenons pas votre refus d'indexer la SCSP sur le volume de repas fournis. Enfin, puisque je suis le dernier

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, madame la rapporteure spéciale, monsieur le rapporteur spécial, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la qualité de vos interventions et de vos remarques.

supplémentaires pour l'Ipev. Une telle augmentation est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte économique compliqué, alors que le Gouvernement engage des dépenses massives en faveur de la préservation du pouvoir d'achat des Français, qui est bien sûr notre priorité. Les crédits alloués au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 2023 s'élèvent ainsi à 25,7 milliards d'euros, répartis entre les trois programmes, 150, 172 et 231, qui relèvent de ma responsabilité. La Mires rassemble également des programmes relevant d'autres ministères : le programme 190 relève du ministère de la transition écologique, le programme 191 du ministère des armées,

Ce programme a pour finalité d'assurer à la France, et à l'Europe l'ESA, la maîtrise des technologies spatiales nécessaires pour progresser dans la connaissance de l'univers, pour mieux quantifier l'impact du changement climatique sur notre planète et pour garantir notre autonomie stratégique sur les enjeux de souveraineté. Le projet de loi de finances pour 2023 illustre cette ambition renouvelée, soulignée par la Première ministre voilà quelques semaines devant le Congrès international d'astronautique.

Le budget pour 2023 porte également la compensation aux établissements d'enseignement supérieur, aux organismes de recherche et au Cnous de la revalorisation du point d'indice des agents publics

: 114 millions d'euros supplémentaires destinés à améliorer la rémunération et les carrières de l'ensemble des personnels. Ces revalorisations et requalifications d'emplois concernent l'ensemble des agents, fonctionnaires ou contractuels, sous statut de droit public ou privé, travaillant dans des organismes de recherche ou dans des universités. Je souligne- c'est important -que la hausse du point d'indice s'ajoute à ces mesures : elle ne s'y substitue pas.

la LPR ne prévoyait pas de montée en charge pour 2023. On peut déjà souligner les effets visibles de l'augmentation de l'enveloppe d'engagement, qui a permis- c'était l'objectif -de porter le taux de sélection des projets à hauteur En crédits de paiement, la montée en charge des projets sélectionnés se traduit logiquement par une hausse d'environ 44 millions d'euros. En troisième lieu, une somme de 91 millions d'euros est prévue pour rehausser les budgets des organismes de recherche et des universités, afin de garantir la soutenabilité de leur recrutement, mais aussi d'augmenter la dotation de base aux laboratoires. En quatrième lieu, d'autres augmentations, pour un montant total de 81 millions d'euros, permettre d'investir dans les grands équipements scientifiques et de renforcer le lien entre la science et la société la diffusion de la culture scientifique et le transfert des résultats de la recherche vers le monde des entreprises. Enfin, les 650 créations de postes prévues par la LPR viendront soutenir l'attractivité de la recherche, avec 179 nouvelles chaires de professeur junior, 377 contrats doctoraux supplémentaires et 94 postes de titulaires dans les organismes de recherche. Vous le voyez, le budget pour 2023 traduit mon engagement de réinvestir dans la recherche en poursuivant la dynamique de la LPR, sans rien enlever à notre ambition commune.

Le deuxième bloc renvoie aux 364 millions d'euros prévus pour la compensation de la revalorisation du point d'indice. Quant au troisième bloc, sur lequel je vais dire quelques mots plus précis, il regroupe environ 160 millions d'euros de mesures nouvelles en faveur de l'enseignement supérieur.

est soumis est la traduction budgétaire des mesures majeures annoncées avant l'été par le Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat de tous nos étudiants. Je citerai les deux principales, qui

intégralement compensé par l'État. Le PLF pour 2023 permet également de renforcer l'accompagnement des étudiants, de mieux protéger leur santé, de mieux prendre en compte leurs difficultés. Je pense au doublement des moyens consacrés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, soit une hausse de 7,5 millions d'euros, conformément aux conclusions du comité interministériel au handicap de février 2022.

Ces services devront s'ouvrir à l'ensemble des étudiants et se rendre plus accessibles. Les crédits ouverts l'an dernier pour financer l'ouverture de 80 postes de psychologues et la distribution gratuite de protections périodiques sont par ailleurs pérennisés.

Avant de conclure, je voudrais rappeler qu'au budget du ministère s'ajoutent les crédits de France 2030. La recherche et l'innovation sont à la source des nouvelles découvertes, qu'il s'agisse des fonds marins ou de l'espace, de nouveaux médicaments ou du nucléaire, d'agriculture ou de mobilités propres. Le déploiement de ces innovations nécessitera de former de nouveaux talents, en s'appuyant, entre autres, sur l'excellence de nos sites universitaires et de tous nos établissements. Ainsi, plus de 13 milliards d'euros seront investis bénéfice des acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation sur la période 2020-2027, qui verra l'ouverture de places supplémentaires pour des formations nouvelles.

Cela traduit l'engagement renouvelé du Gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, en faveur de nos étudiantes et de nos étudiants, donc en faveur de notre avenir. Nous allons

Si des programmes exceptionnels ont bien été mis en oeuvre à la faveur des crises, ils ne répondent pas au besoin global de financement de l'immobilier universitaire, ce financement demeurant profondément défaillant. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur estime à 7 milliards d'euros le coût des réhabilitations en attente, liées aux exigences de la transition énergétique et environnementale. Pour sa part, France Universités retient un montant de 15 milliards d'euros pour une rénovation totale.

la crise sanitaire n'a rien arrangé : sédentarité, cours à distance, augmentation du temps passé devant les écrans. Cette baisse de l'activité physique représente un facteur de risque important pour la santé mentale, physique et sociale des étudiants. Il est donc urgent de renforcer la place du sport à l'université, y compris dans le cursus universitaire de chaque étudiant. Mais cela n'est réalisable qu'à la condition que chaque université soit dotée d'infrastructures sportives de qualité et accessibles à tous.

Lors de la crise sanitaire, le Gouvernement a annoncé l'extension des repas à un euro à tous les étudiants, boursiers et non boursiers. Malheureusement, cette mesure a été supprimée à la rentrée universitaire 2021, le repas à un euro étant de nouveau réservé aux seuls étudiants boursiers. Pourtant, la précarité étudiante ne cesse de progresser dans notre pays. D'après la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), 62 % des étudiants ont des difficultés pour se nourrir correctement. De nombreuses associations organisent régulièrement des distributions alimentaires ; le Gouvernement a d'ailleurs débloqué 10 millions d'euros pour soutenir leur action. C'est bien, mais nous attendons des réponses plus structurelles

Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 20 % des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 46 % d'entre eux exercent au moins une activité salariée durant leurs études.

La majorité des étudiants boursiers bénéficient des bourses sur critères sociaux dix mois par an et ne perçoivent plus rien en juillet et en août. Pourtant, vous le savez, le loyer et les charges de la vie courante ne s'arrêtent pas en juin. Selon une enquête menée par Diplomeo, 70 % des étudiants travaillent en juillet et en août et 53 % d'entre eux sont obligés de travailler pour financer leurs études. En outre, ils sont de plus en plus nombreux à faire des stages ou à étudier durant la pause estivale

Cette mesure est loin d'être superflue, à l'heure où 20 % des étudiants français vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cet amendement vise à financer le surcoût de l'énergie pour les universités, dans le contexte exceptionnel que nous connaissons. L'actualité a montré que ce surcoût pourrait se traduire par la fermeture temporaire de certaines universités. Or il paraît inconcevable que la vie universitaire s'en trouve affectée et que ce coût soit indirectement supporté par les étudiants, qui se retrouveraient de nouveau en distanciel, chez eux, dans des logements que l'on sait précaires et avec des factures d'électricité qui explosent. Ainsi, par cet amendement, nous demandons que l'État double la rallonge budgétaire

entre janvier et septembre 2021, l'extension des repas à un euro aux étudiants non boursiers a permis de multiplier par cinq le nombre de repas distribués chaque semaine : près de 178 000 étudiants non boursiers ont pu bénéficier d'au moins un repas pendant cette période, contre moins de 50 000 habituellement. Les chiffres sont éloquents, alors même qu'à cette période les étudiants n'étaient pas de retour à temps plein sur les campus. En pleine période inflationniste et alors que sévit la crise énergétique, il est essentiel de rétablir cette aide quotidienne à destination de tous les étudiants précaires

dont la santé physique et mentale a été gravement affectée par la pandémie et par la hausse du coût de la vie, en déployant une offre complète de prévention et de soins sur l'ensemble du territoire. Il est devenu urgent de faire de la santé étudiante une priorité. une priorité. Selon la Fage, 40 % des étudiants ont renoncé à se soigner depuis le début de la crise du covid-19, en mars 2020. Parmi eux, 43 % l'ont fait pour des raisons financières,

Mme Monique de Marco. Dans notre pays, plus de 990 000 étudiants renoncent à des soins par manque de moyens. En effet, si la sécurité sociale rembourse environ 70 % des dépenses les 30 % restants représentent une somme significative dans le budget d'un étudiant. Cette réalité est d'autant plus forte que 36 % des étudiants ne sont pas couverts par une complémentaire santé, principalement par manque de moyens. Selon l'Union nationale des étudiants de France (Unef), le coût de la santé atteint 134 134 euros par an dans le budget d'un étudiant sans complémentaire. De surcroît, ce coût augmente chaque année avec l'inflation, contrairement aux aides perçues par les étudiants.

Bernard Fialaire. Cet amendement tend à relever le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig), fixé à 94,9 millions d'euros dans la mission « Recherche et enseignement supérieur

représente au total près de 160 000 étudiants supplémentaires. L'augmentation des effectifs étudiants en formation initiale dans ces établissements ne s'est pas accompagnée de l'effort budgétaire correspondant. d'étudiants, les subventions publiques octroyées par l'État aux établissements privés labellisés d'intérêt général ont donc baissé drastiquement : elles ont été divisées par deux en dix ans et ne représentent plus que 596 euros par étudiant, soit un vingtième du coût moyen de la formation.

qui pourraient d'ores et déjà être mobilisés par les différents partenaires, déterminer la gouvernance du projet et enfin mobiliser les équipes sur le sujet. » En gras, dans le même rapport, on trouve aussi cette information assez inattendue : « L'Inserm a indiqué au rapporteur spécial qu'à ce stade des financements supplémentaires inscrits en loi de finances n'étaient pas nécessaires Or, selon les associations de patients, rien n'indique qu'un programme concret de recherche soit en train d'émerger et que des financements aient été trouvés. Cette situation nous interpelle

dernière est essentielle à la transition énergétique, agricole et industrielle que nous menons. Cet amendement vise à renforcer les moyens alloués à la recherche dans le domaine environnemental : je vous propose de réorienter 20 millions d'euros du programme « Recherche spatiale » vers ce secteur déterminant pour notre avenir. L'importance de la recherche spatiale n'est plus à démontrer, mais son budget augmente déjà de 223 millions d'euros. du climat (Giec) est clair : nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prendrons et les investissements que nous réaliserons peuvent nous garantir un avenir vivable. Pourtant, alors même que le Gouvernement défend les mérites de l'innovation et qu'il augmente le budget de la recherche spatiale de 223 millions d'euros, les moyens alloués à la recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement baissent de 0,5 % en 2023. La construction et les transports

Marco. Alors que 33 % des étudiants renoncent à des soins par manque de moyens, il est nécessaire de renforcer l'offre des services de santé universitaire et interuniversitaire. Cet amendement vise à augmenter de 3 millions d'euros les moyens attribués à ces services afin qu'ils puissent remplir leur mission de service public. Éléments clés du parcours de santé des étudiants, ils sont essentiels en matière de prévention, de contraception, de suivi vaccinal et d'accompagnement psychologique

présent PLF. Les étudiants boursiers pourront aussi solliciter l'attribution d'un Pass'Sport à hauteur de 50 euros par an. J'émets, partant, un avis défavorable

Je partage la préoccupation des auteurs de l'amendement n° II-520 : la santé des étudiants est une question cruciale dans le contexte actuel. Je suis donc favorable à la mise en place d'un accompagnement plus personnalisé. En revanche, je doute du caractère opérationnel de l'amendement

recourir à l'emprunt ou à des montages innovants, comme le tiers financement, et mobiliser les capacités financières des établissements lorsque ces derniers ont déjà prévu

par an- ces éléments sont sans doute à l'origine des précisions contenues dans le rapport de M. le député Bouloux. Dans ce cadre et à la demande du ministère de la santé et de la prévention,

et l'accessibilité du bâti feront partie des huit domaines prioritaires de la prochaine Conférence nationale du handicap, qui se tiendra au printemps prochain et qui sera l'occasion de mettre en oeuvre de nouvelles actions concrètes. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement engagé

dans laquelle sont notamment investis l'Institut pour la recherche en santé publique et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le handicap est progressivement devenu un enjeu majeur des politiques publiques. Cependant, les retards accumulés nécessitent une mobilisation importante

sénateurs, vous le voyez, le Gouvernement soutient avec conviction la recherche sur le handicap et les acteurs qui la conduisent. Ces projets de recherche doivent être menés dans le cadre d'une concertation permettant de définir des actions

Enseignement supérieur et recherche agricoles », et de minorer de ce même montant l'action n° 05, Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique, du programme 193 « Recherche spatiale

défendu. Quel est l'avis de la commission ?

ou aux opérateurs publics qui le souhaitent, afin de leur permettre de développer une offre de restauration au bénéfice- non nécessairement exclusif - des étudiants, et ce à des tarifs adaptés.

Toutefois, la commission a un doute sur le rattachement de cet amendement au domaine des lois de finances. Avis de sagesse.